La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

venue rencontrer plusieurs de nos collègues dans le cadre de l’examen du projet de loi d’urgence pour Mayotte, adopté à l’unanimité par

Je souhaite leur témoigner, au nom du Sénat, toute notre sympathie. Nous savons combien ils ont été sollicités par la population qui était – et reste – en état de détresse après le passage du cyclone Chido. Je veux les assurer de notre pleine solidarité. Le Sénat a veillé, au cours de ses travaux, à enrichir le projet de loi d’urgence qui lui était soumis en vue non seulement de reconstruire plus vite, mais aussi et surtout de reconstruire mieux. Il a également souhaité garantir l’association des élus mahorais

L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement. J’excuse l’absence de M. le Premier ministre, qui est retenu à l’Assemblée nationale pour la discussion et le vote de deux motions de censure.

Monsieur le ministre, qui gouverne réellement la France ? L’État et ses élus ou les multinationales et leurs lobbys ? L’affaire Nestlé est en train de devenir un terrible scandale d’État. Les révélations de l’enquête menée par Radio France et sur Nestlé confirment en tout point ce que je dénonçais, en octobre 2024,

Hier, nous apprenions de surcroît que Nestlé a fraudé au vu et au su de l’Élysée ! Depuis 2017, Emmanuel Macron offre liberté et largesses aux multinationales. Je ne m’étendrai pas sur les Uber Files – vous savez parfaitement de quoi je parle… Je dénonce ici le rapport plus que problématique de la Macronie avec les intérêts privés.

ils leurs emplois. Pourquoi l’Élysée et Matignon ont ils autorisé Nestlé Waters à frauder au mépris de la sécurité sanitaire et de la réglementation européenne ? Comment pouvez vous justifier que cette fraude perdure ?

tous les documents qui ont été demandés ont été transmis. Sachez que mon ministère est pleinement engagé pour faire toute la transparence sur la qualité de l’eau embouteillée,

Monsieur le ministre, à l’issue d’un débat constructif, le Sénat a adopté à l’unanimité le projet de loi d’urgence pour Mayotte. Dès l’article 1, nous avons inscrit dans le texte le rôle incontournable des collectivités territoriales le président du conseil départemental, les communes et les intercommunalités – dans le pilotage de l’établissement chargé de la reconstruction de l’archipel. Je salue à mon tour les présidents d’intercommunalité mahorais présents aujourd’hui dans les tribunes Pour que la reconstruction soit durable, l’adaptation à la réalité locale est un enjeu primordial, qui exige une coconstruction étroite avec les collectivités locales.

Je tiens à saluer à mon tour la présence de quatre présidents d’intercommunalités mahoraises à Paris cette semaine. Je voudrais leur dire, au nom du ministre d’État, ministre des outre mer, Manuel Valls, qu’ils seront reçus demain au ministère des outre mer et que la porte de la rue Oudinot leur sera toujours ouverte. La semaine dernière, le ministre d’État, ministre des outre mer a signé avec le président du conseil départemental et le président de l’association des maires de Mayotte une convention d’intention posant les principes qui doivent guider la reconstruction et la refondation de Mayotte. Je réaffirme devant vous un principe clair, qui vient d’être mentionné par le président du Sénat : il n’y aura pas de reconstruction ni de refondation de Mayotte sans une coopération étroite, je tiens à le dire, entre l’État et les collectivités territoriales mahoraises. Que ce soit en matière de développement économique, d’environnement, de cohésion sociale ou d’urbanisme, le retour d’expérience des communes et des intercommunalités sera essentiel pour préparer la reconstruction et élaborer la loi programme. Je veux également vous dire, sans préjuger des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d’urgence, que l’article 1dudit texte prévoit, dans sa rédaction actuelle, « une représentation équilibrée des représentants de l’État et des collectivités territoriales de Mayotte

Aucune projection dans l’avenir, vous le savez, ne sera possible sans le rétablissement de la sécurité, qui passe par la régulation migratoire.

pour migrants sans papiers, traitements dégradants imposés à des personnes lors de leur expulsion vers leur pays d’origine, recul spectaculaire des droits des minorités,… Encore bravo ! … guerre commerciale mettant en péril l’économie mondiale, menace d’imposer des droits de douane sur les produits se pourrait que cette liste à la Prévert continue longtemps de s’allonger, tant le président américain a été proactif dans la mise en œuvre de politiques consternantes depuis son retour aux affaires. sortie en date, il a déclaré la nuit dernière sa volonté de prendre le contrôle de la bande de Gaza pour en faire la « Côte d’Azur du Moyen Orient », au mépris absolu du droit international et de la sécurité des otages. On ne peut en effet appréhender On ne peut en effet appréhender qu’avec inquiétude les conséquences des politiques de Donald Trump, lequel entraîne dans son sillage les grands patrons américains qui contrôlent les principales sources privées d’influence aux États Unis. Je prendrai pour exemple les nouvelles « règles de la communauté » qui autorisent désormais à tenir des propos haineux, ainsi que la suppression du programme de des contenus publiés sur lesdits réseaux, porte ouverte à la désinformation. décision a été saluée par Elon Musk, qui utilise son propre réseau social, X, pour s’ingérer dans les processus électoraux et démocratiques européens. Je rentre des États Unis, où l’on m’a déjà fait part d’ingérences, y compris dans nos établissements du réseau d’enseignement français à l’étranger, à l’étranger, par l’instauration d’un climat délétère et la remise en question de certaines de nos valeurs fondamentales. Ma question est simple, monsieur le ministre : comment la France compte t elle peser au sein de l’Union européenne afin de s’affirmer comme la puissance stratégique qu’elle doit être face à un allié qui se fait de plus en plus menaçant ? La

à la multiplication des annonces tous azimuts outre Atlantique, il nous faut évidemment garder notre sang froid et rappeler ce que nous sommes et ce que nous voulons.

qui serait une atteinte aux aspirations légitimes du peuple palestinien et qui entraverait la mise en œuvre d’une solution à deux États, seule susceptible d’apporter la paix et la stabilité dans la région.

sans aucune espèce d’hésitation. Pour ce qui concerne les géants du numérique, l’Europe s’est donné des règles. Elle refuse que le débat public soit délocalisé sur des plateformes de réseaux sociaux dont les règles seraient fixées par des milliardaires américains ou chinois. Là encore, si ces règles sont transgressées – des enquêtes sont en cours –, les plateformes doivent être sanctionnées lourdement par la Commission européenne, qui peut prononcer des amendes allant jusqu’à 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial de la société concernée et pousser les sanctions jusqu’à la restriction d’accès sur le territoire de l’Union européenne. Que fait la France pour peser dans ce débat ? Le Président de la République a participé lundi dernier à une retraite des chefs d’État et de gouvernement embrassant l’ensemble de ces sujets. Quant à moi, je réunirai le 12 février prochain les principaux pays européens afin que nous abordions la « suite des opérations », si je puis dire, autour d’un discours uni, ferme et serein face à ce qui peut arriver ou ce qui peut provenir des États Unis d’Amérique dans un avenir prochain. La parole est à Mme Marie Claude Lermytte, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Depuis 2010, ces crèches, qu’elles soient privées ou publiques, se sont développées grâce à la souplesse dont elles bénéficient en matière d’encadrement. Elles ont en partie comblé un manque, notamment en milieu rural, où l’offre d’accueil de la petite enfance reste insatisfaisante. Rappelons à cet égard qu’un enfant sur trois vit dans une commune rurale. Aujourd’hui, les microcrèches représentent 13 % de l’offre totale : le soutien qu’elles apportent est donc essentiel. Leur succès est indéniable, mais leur avenir semble menacé. En imposant des contraintes trop abruptes, ce décret risque de provoquer une vague de fermetures. Sachant qu’il manque déjà 10 000 professionnels dans le secteur de la petite enfance, peut on vraiment se permettre de perdre un grand nombre de places d’accueil d’ici à 2026 ? Soyons clairs : il ne s’agit pas de remettre en cause l’alignement des exigences en matière de diplôme. Un enfant est un enfant, quel que soit son mode d’accueil ou son lieu de vie.

Bien que vous mettiez l’accent sur la priorité donnée aux métiers en tension, il est crucial de rappeler que certains secteurs essentiels pour le fonctionnement de nos entreprises font face à un manque de main d’œuvre structurel.

Le recours à des médecins étrangers nous permet par exemple de pallier le problème des déserts médicaux. En durcissant les critères d’intégration, vous risquez de priver de nombreuses entreprises françaises de ressources humaines indispensables à leur activité, tout en mettant en difficulté les personnes étrangères qui, à défaut de régularisation, se trouvent dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins. Voilà qui pourrait aggraver la précarisation de ces personnes et engendrer un risque accru de recours au travail dissimulé et de développement des trafics. L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) s’inquiète de l’impact de cette circulaire sur les conditions de régularisation et d’accès à l’emploi, et demande expressément que les mesures prises ne durcissent pas les critères applicables aux ressortissants étrangers déjà présents sur notre sol et désireux de travailler dans des métiers en tension. Ladite circulaire risque non seulement d’aggraver la pénurie de main d’œuvre dans ces secteurs cruciaux, mais aussi de compromettre le respect de la dignité et des droits des travailleurs étrangers qui contribuent, souvent dans des conditions précaires, au bon fonctionnement de nos entreprises et à la croissance économique du pays. Dans ce contexte, monsieur le ministre,

c’est une question pertinente que vous posez. Autant nous devons être d’une fermeté exemplaire à l’égard des étrangers en situation irrégulière, qui doivent être reconduits dans dans leur pays d’origine, autant, en matière d’immigration, nous devons réorienter nos choix. Je partage l’idée selon laquelle l’immigration économique qualifiée doit être une priorité : le Gouvernement y travaille. Très bien

plus de 4 millions de Français sont mal logés et, parmi ceux qui ont un toit, 30 % indiquent avoir eu froid dans leur logement l’an passé. Ces constats sont ceux de la Fondation pour le logement des défavorisés, qui présentait hier son trentième rapport sur l’état du mal logement en France. Oui, cela fait huit ans qu’année après année notre pays s’enfonce toujours un peu plus dans la crise du logement, les réponses des gouvernements successifs étant loin d’être à la hauteur. Pour nombre de nos compatriotes qui cherchent à se loger, particulièrement les plus modestes, c’est tout simplement un parcours du combattant La situation est inédite : durcissement de la crise de la construction, grippage du marché immobilier, effets de l’inflation, aggravation des inégalités… Les files d’attente s’allongent pour obtenir un HLM. À la fin du mois de juin, l’Union sociale pour l’habitat (USH) recensait 2,7 millions de ménages demandeurs. Là encore, les chiffres sont à la hausse, d’autant plus que la production de logements sociaux est au plus bas depuis vingt ans. Comment pourrait il en être autrement ? L’effort public en faveur du logement est tombé à 1,5 % du PIB, son plus bas niveau depuis trente Faute d’être reconnu comme une priorité, le logement a été délaissé. De fait, 2024 aura été une nouvelle année de renoncement. Madame la ministre, allez vous enfin agir pour résorber le mal logement ?

Le crash de l’application Lucie est le terrible exemple d’une industrie détricotée et d’une recherche affaiblie, une nouvelle fois amputée, dans votre budget, La question est pourtant existentielle : la France sera t elle vassalisée par ces nouveaux impérialismes, ou sera t elle capable de bâtir une régulation plus ambitieuse que l’européen, bien trop timoré, face aux tyrans numériques ? L’IA doit être un bien commun de l’humanité, mis au service de progrès humains, écologiques et scientifiques, et non un outil détenu par quelques milliardaires et mis au service de leurs seuls profits. À cet égard, votre politique du « en même temps » est intenable dénoncer – à raison – l’alliance internationale de tous les réactionnaires et en même temps dérouler le tapis rouge à Elon Musk, l’homme qui fait des saluts nazis et s’invite au congrès de l’AfD () après avoir participé à la victoire de Trump met sa fortune au service de la désinformation – X –, des guerres commerciales et des conquêtes coloniales, du Groenland à Gaza, contribuant à accélérer encore la destruction de l’ensemble du vivant ! Madame la ministre chargée de Gouvernement de signifier clairement à Elon Musk qu’il n’est pas le bienvenu à ce sommet, car nous ne partageons pas son projet de société ; d’agir pour le développement d’une IA éthique, fiable et souveraine à l’échelle européenne ; et de proposer une COP mondiale sur l’IA sous l’égide des Nations unies. Bravo ! La parole

c’est que nous sommes au début de cette technologie et que la meilleure réponse est la nôtre : investir – investir dans nos talents,… Trop tard ! … les chercheurs français étant reconnus dans le monde entier, investir dans nos infrastructures

voilà vingt ans, nous nous étions assis tous ensemble pour développer les technologies du numérique, nous n’en serions pas là aujourd’hui. La meilleure réponse

Madame la ministre, notre département a été frappé par des crues historiques : Rennes, Guipry Messac, Redon, Bruz, Guichen, Pacé, Noyal Châtillon sur Seiche autant de communes dont les habitants ont affronté la montée des eaux de l’Ille, de la Vilaine et de la Seiche alors qu’à la dépression Herminia a succédé la tempête Éowyn. Face à cette situation inédite pour notre territoire,

mais également aux forces de sécurité et de secours – les pompiers, la sécurité civile, les services de la préfecture –, qui continuent en ce moment même d’œuvrer pour protéger les populations et répondre à l’urgence.

Ces événements s’inscrivent dans le cadre du changement climatique, qui démultiplie et augmente l’intensité des épisodes extrêmes. Face à ces risques accrus, les communes sont de plus en plus confrontées à des refus d’assurance.

Tous ont tiré la sonnette d’alarme sur les difficultés croissantes que rencontrent les collectivités pour obtenir une couverture d’assurance. Madame la ministre, nos élus ont engagé leurs communes, leurs services et les budgets communaux pour pallier l’urgence.

individus sont dehors. Reconnaissez qu’on est chez les fous… Monsieur le garde des sceaux, nous connaissons votre détermination et celle du ministre de l’intérieur à lutter contre le narcotrafic. Nous avons voté hier à l’unanimité un texte important pour nous donner les moyens de mener ce combat. Votre question ! Qu’allez vous faire pour répondre à cette folie procédurière, qui décourage nos policiers et nourrit la colère et l’incompréhension de nos concitoyens ? La parole

le problème que vous soulevez traduit la complexité de la procédure en matière de droit des étrangers, et singulièrement lorsque ceux ci sont placés en centre de rétention.

La parole est à M. Yan Chantrel, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

le pouvoir d’achat et la justice sociale sont les grands oubliés de votre budget pour 2025 : pas de coup de pouce sur le Smic ni de revalorisation de la prime d’activité en faveur des travailleurs modestes, aucune augmentation du point d’indice pour les fonctionnaires, quand 30 % de nos compatriotes n’arrivent pas à boucler leurs fins de mois ! Pendant ce temps, les écarts de rémunération s’accroissent. À la fin de 2024, la famille Mulliez s’est versé 1 milliard d’euros de dividendes grâce aux profits de Décathlon, tout en supprimant 2 400 emplois chez Auchan… Le patron de Carrefour, qui gagne 426 fois plus que la moyenne de ses salariés, est le symbole de l’indécence des écarts de revenus qui perdurent dans notre pays. Pourtant, vous refusez toujours de remettre en place un d’augmenter le taux de la et de taxer les superdividendes ! Quand prendrez vous la mesure de la crise sociale qui sévit dans notre pays ? Quand agirez vous concrètement pour augmenter le pouvoir d’achat de ceux qui n’ont que leur travail pour vivre ?

Je vous donne un cas très concret : lors de l’audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire de Melun, le procureur de la République a annoncé le classement sans suite et sans acte d’investigation d’un certain nombre de plaintes, et ce pour « désengorger » les tribunaux et « alléger le travail des policiers ». Les plaintes seront désormais « triées dès l’origine en fonction des priorités » et le procureur de la République a lui même reconnu que cela était « choquant sur le principe À l’heure où nombre de nos concitoyens n’osent pas porter plainte, y compris pour des faits très graves, le signal que la justice envoie est dévastateur. Celle ci doit être au service des victimes, non des délinquants Tout cela induit une perte de sens pour les juges, pour les policiers, mais aussi pour les citoyens. L’argument du manque de moyens humains et financiers est inaudible

Monsieur le garde des sceaux, nous savons que le ministère de la justice est le ministère du temps long. Nous comptons sur vous pour agir, car les Français ne peuvent plus se contenter d’une justice pour les délinquants ; ils ont besoin d’une justice pour les victimes !

Votre texte doit au contraire être un outil pour nous permettre d’atteindre trois objectifs que nous partageons : premièrement, réaffirmer notre confiance envers les élus locaux et les mettre au cœur du dispositif

pour la réussite de notre ambition collective en matière de sobriété foncière.

La parole est à M. François Bonhomme, pour le groupe Les Républicains.

les actions violentes et les occupations illégales qui entravent le chantier de la LGV Toulouse Bordeaux sont inacceptables et seront traitées avec la plus grande fermeté.

ferroviaires européennes – cette ligne est un maillon essentiel pour relier la péninsule ibérique au reste de l’Europe. Je rappelle que ce projet a fait l’objet de toutes les procédures de concertation nécessaires et qu’il bénéficie de toutes les autorisations légales. Par ailleurs, les collectivités territoriales sont pleinement engagées au côté de l’État, le financement étant partagé. Les opposants ne peuvent pas s’arroger le droit de bloquer un chantier d’utilité publique, attendu par la majorité de nos concitoyens. L’État prendra donc toutes les mesures nécessaires pour garantir la poursuite des travaux, dans le respect du calendrier prévu, tout en assurant, bien sûr, la sécurité de l’ensemble des professionnels intervenant sur le chantier. Je pense notamment aux ouvriers, qui sont trop souvent menacés avec des armes par destination. Quelles que soient les motivations de ces opposants, c’est tout simplement intolérable

selon un scénario immuable, ces faux rebelles, qui montent aux arbres, au sens propre comme au sens figuré, pour contester tout projet, annoncent la sempiternelle « convergence des luttes » avec les opposants à l’A69, entre Castres et Toulouse. Nous ne voulons plus de cette faiblesse chronique ni de ces faux fuyants qui ont si souvent été l’antichambre du renoncement de l’État

La parole est à Mme Marion Canalès, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Faut il que tout change pour que rien ne change ? Sous couvert d’un choc de simplification censé renforcer la compétitivité, la Commission européenne travaille depuis aujourd’hui à faire reculer la lutte contre le réchauffement climatique et pour la défense des droits humains et sociaux. Ce n’est pas une mince affaire… Bien sûr, il

Des organisations patronales professionnelles, des ministres et même des multinationales défendent ces textes. À leur sujet, certains évoquent un moratoire ; mais le moratoire est l’antichambre du renoncement. La France va t elle renoncer à tenir son rôle, en Europe, en faveur de la transition écologique ? Allons nous faire comme si le défi climatique n’était pas un sujet, alors qu’il se rappelle à nous tous les jours À qui rendons nous service en reculant ainsi ?

aujourd’hui. Pour les grandes entreprises, nous proposons un plafonnement du dans la chaîne de sous traitance et un alignement sur les obligations simplifiées applicables aux PME cotées.

Madame la ministre, le pouvoir d’achat reste de loin la principale préoccupation des Français. Nous assistons à un phénomène dont on parle peu, mais qui prend de l’ampleur dans notre pays : beaucoup de Français ne font que survivre, alors même qu’ils travaillent. ces travailleurs pauvres est en constante augmentation. Je parle bien de travailleurs, car il s’agit en grande partie de gens qui se lèvent tôt, à trois ou quatre pour exercer des tâches pénibles. Ce sont des courageux et de vrais productifs : principalement des ouvriers dans les usines et les ateliers, des agriculteurs, des salariés de la restauration et de l’entretien.

C’est pourquoi nous devons continuer à soutenir les négociations sur les salaires au niveau des branches et des entreprises. La semaine dernière, j’ai réuni le comité de suivi des salaires, qui regroupe l’ensemble des partenaires sociaux à l’échelle nationale, pour faire le point sur l’état des minima de branche. Les branches jouent le jeu, à l’exception de cinq d’entre elles, pour lesquelles les négociations sont durablement bloquées. Trois

La place d’une femme est à la demeure auprès de son père. Crains ton Seigneur » : ce propos n’est pas une citation d’un théoricien d’Al Qaïda ; il émane de la nouvelle recrue de l’émission star de France 5,, qui réunit un million de téléspectateurs en moyenne chaque soir. Cet humoriste

La polémique suscitée par son intronisation sur France 5 l’a conduit à fermer ses réseaux au public et à les nettoyer… au kärcher. J’ajoute que cet « humoriste » annonce la couleur, avec son look salafiste. Si l’habit ne fait pas le moine, reconnaissons que le propos fait le salafiste. Comment peut on participer, avec l’argent du contribuable, à normaliser les idées que véhicule ce personnage ? Est ce bien ce que l’on attend du service public de l’audiovisuel et de ses maisons de production ?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

L’ordre du jour appelle la désignation des vingt trois membres de la commission d’enquête sur les missions des agences, opérateurs et organismes consultatifs de l’État. En application de l’article 8, alinéa 5 de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées.

de la mer – FranceAgriMer – accompagne les interprofessions et les filières afin qu’elles définissent une stratégie assortie d’objectifs, notamment de production, à horizon de dix ans,

parmi les priorités des politiques en faveur de la souveraineté alimentaire, en lien avec le renouvellement des générations d’actifs. Aux termes de l’article 1,

vise à réintroduire de manière concise les enjeux d’alimentation de la population dans les priorités de notre politique en faveur de la souveraineté alimentaire. « Assurer à l’ensemble de la population, dans le cadre

On ne peut pas laisser au seul secteur privé le soin de définir une politique alimentaire. Ce n’est pas sa vocation ; en revanche, c’est celle de l’État.

texte qui mentionne l’alimentation. Toutefois, il supprime la notion même de politique de l’alimentation et réduit le périmètre des actions à mener, dans un rôle unique de maintien et de développement des filières. Cela n’est pas suffisant.

mais ne consommons que 63 % de fruits tempérés produits en France. Nous exportons donc le quart de notre production de fruits tempérés, pour importer 37 % de ceux que nous consommons.

La souveraineté alimentaire consiste fondamentalement à produire en France ce que l’on consomme en France. Si des filières ne sont pas rentables, il revient à la puissance publique de les accompagner pour garantir notre souveraineté et non aux marchés mondiaux d’imposer leurs règles. Le secteur agricole est mis à mal par l’ouverture croissante au libre échange, bafouant, de surcroît, les problématiques sociales et environnementales. Préciser la nécessaire corrélation entre la production nationale et les besoins alimentaires de la population

remplacer la notion de compétitivité par l’objectif d’un haut niveau de performance qualitative, sanitaire, environnementale et sociale. Je partage tous ces objectifs. Pour autant, pourquoi éliminer, singulièrement, la dimension économique des exploitations ?

l’agriculture française.

L’objectif d’une agriculture économiquement et écologiquement viable, rémunératrice, diversifiée, durable, répartie sur l’ensemble du territoire et capable de produire une alimentation saine, sûre, nutritive et accessible à tous, conformément au principe de souveraineté alimentaire, doit prédominer et servir de mise en garde contre l’opposition stérile entre agriculteurs et environnement. C’est pourquoi cet amendement tend à rappeler que la recherche et l’innovation ne peuvent, à elles seules, répondre aux défis engendrés par le changement climatique. Il vise ainsi à consacrer l’adaptation de l’agriculture au changement climatique comme une priorité majeure de la politique en faveur de la souveraineté alimentaire. L’accompagnement du monde agricole face à ce défi climatique sera essentiel pour continuer à produire sur notre territoire dans les années à venir.

nécessaire d’accompagner les agriculteurs, y compris en soutenant la recherche et l’innovation, et de surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte aux capacités de production nationale et à l’approvisionnement alimentaire. La parole à rappeler que la recherche et l’innovation ne peuvent, à elles seules, répondre aux défis engendrés par le changement climatique. Il vise ainsi à consacrer l’adaptation de l’agriculture au changement climatique comme une priorité majeure de la politique en faveur de la souveraineté alimentaire. L’accompagnement du monde agricole face à ce défi climatique sera essentiel pour continuer à produire sur notre territoire dans les années à venir.

De rechercher des solutions techniques et scientifiques d’adaptation au changement climatique et d’accompagner les agriculteurs pour surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte aux capacités de production

Pourtant, sans foncier agricole accessible et disponible, sans une lutte accrue contre la spéculation foncière, la France ne pourra pas relever le défi du renouvellement des générations. Sans ce renouvellement des générations, nous ne préserverons pas

de l’article 8 est en effet ainsi rédigé : « Pour atteindre cette cible, l’État se fixe pour objectif de contrôler les phénomènes d’agrandissement par la régulation de l’ensemble des marchés fonciers afin de permettre le renouvellement des générations en agriculture. La réalisation de cet objectif suppose de préserver les terres agricoles, de rendre le foncier accessible aux candidats à l’installation et de faciliter la transmission des exploitations agricoles. À cette fin, une réforme de l’ensemble des instruments juridiques et financiers doit permettre à la politique foncière de s’adapter aux enjeux contemporains.

proposition de M. le rapporteur invite la France à se placer en queue de peloton de l’Union européenne en matière de normes sociales et environnementales. Loin de moi l’idée de faire injure à certains de nos voisins européens, mais il n’est dans l’intérêt ni de nos agriculteurs, ni des travailleurs agricoles, ni de notre environnement, ni même de nos paysages, d’abaisser nos exigences au niveau des plus mauvais élèves de l’UE. Nous ne pouvons croire que cette vision capitaliste sans vergogne soit celle de M. le rapporteur, attaché, nous en sommes persuadés, à l’excellence de notre agriculture. Nous regrettons également cette vision souverainiste qui considère que la France doit tirer plus de profit du projet européen qu’elle n’y contribue. Elle n’est pas à la hauteur du rôle historique de notre pays, fondateur

au delà de sa dimension de revenu direct. Pourtant, son fonctionnement actuel ne répond ni au défi de l’installation des jeunes, ni à l’exigence de souveraineté alimentaire, ni à l’urgence de la transition écologique, qui sont trois défis majeurs auxquels notre modèle agricole est confronté. Nos agriculteurs font face à une PAC mal répartie, au détriment des plus petites exploitations, notamment de polyculture et d’élevage, qui sont pourtant essentielles à la vitalité de nombreux territoires. cet amendement, nous proposons une réforme de fond : une meilleure redistribution des aides, un basculement des subventions vers des contrats de transition écologique et une régulation des marchés agricoles pour garantir des prix plus justes. Dans l’immédiat, nous demandons un renforcement massif des moyens alloués aux mesures agroenvironnementales et climatiques (Maec), aux paiements redistributifs et aux aides à l’installation. Nous considérons que le temps est venu d’une PAC plus juste, plus durable et plus cohérente avec l’avenir auquel nous aspirons pour notre agriculture et notre société.

Cette rédaction ouvre la voie à des interprétations beaucoup trop larges et pourrait tirer notre agriculture vers le bas plutôt que vers le haut. Nous avons pourtant, à plusieurs reprises dans le passé, partagé avec la droite sénatoriale la volonté de lutter contre la concurrence déloyale et l’importation de produits ne respectant pas les mêmes normes que les Nous sommes favorables à l’instauration de véritables clauses miroirs et les débats qui ont entouré la question de la signature de certains accords de libre échange démontrent que nous pouvons tomber d’accord sur certaines approches

la possibilité pour la France d’être mieux disante que la réglementation européenne ou d’être plus en avance que ses partenaires européens sur certains sujets, particulièrement environnementaux ou sociaux. Nous entendons souvent dans cet hémicycle que la lourdeur administrative est l’ennemie de nos politiques publiques et, en l’occurrence, de notre agriculture. Or vous nous proposez ici que chaque décision, dès lors qu’elle ne serait pas minimale, soit obligatoirement accompagnée et motivée par une évaluation. Vous entendez donc créer la lourdeur administrative que vous dénoncez par ailleurs. En conséquence, nous proposons la suppression de l’alinéa 13.

à considérer que les autres pays de l’Union européenne seraient indifférents à la santé de leurs populations et que notre pays serait le seul à y être attentif

Afin d’atteindre les objectifs fixés par ce projet de loi, nous devons garantir l’accès à une formation publique gratuite de qualité pour toutes et tous et partout sur le territoire. Il n’y aura pas de renouvellement de générations d’actifs sans formation, pas plus que de transition de l’agriculture ou de maintien de la compétitivité sans enseignement agricole de qualité. Pourtant, la situation de l’enseignement agricole public est critique. Les fermetures des classes et les suppressions de postes se multiplient dans nos territoires. Chez moi, en Nouvelle Aquitaine, ce sont 5 500 heures d’enseignement agricole public qui vont être supprimées. Permettez moi d’évoquer les lycées de

de « favoriser la diversification des profils des porteurs de projets à l’installation », d’« orienter en priorité l’installation en agriculture vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté alimentaire et les transitions écologique et climatique » et de « faciliter l’accès au foncier agricole ». La parole est à

Par cet amendement, il est proposé de traduire la priorité visant à assurer la pérennité et l’attractivité de l’agriculture, ainsi que le renouvellement de ses générations d’actifs par des politiques publiques concrètes englobant l’orientation, l’information, la transmission et l’installation.

également traduire l’engagement de l’État de préserver l’agriculture française en soutenant les jeunes générations, qui en sont l’avenir. Le renouvellement des générations est également menacé par des facteurs structurels, comme les difficultés d’accès au foncier, le niveau d’investissements financiers à consentir ou le manque d’attractivité du métier. À terme, tout cela met en péril non seulement la viabilité de nos exploitations agricoles, mais aussi la sécurité alimentaire, la transition écologique et le maintien de la vitalité de nos territoires ruraux.

Le renouvellement des générations est vital pour assurer la sécurité et la qualité de notre alimentation, produire de la valeur ajoutée économique et environnementale dans l’agriculture et aménager l’ensemble du territoire. Il est à l’origine même de ce projet de loi. Il doit donc être inscrit au sein de cet article programmatique, comme c’était le cas dans la version initiale. Nous ne comprenons pas bien pourquoi une telle

De telles orientations, fondées sur une analyse en silo, favorisent la monoculture, qui est inadaptée à de nombreux terroirs en France.

l’entrepreneur du vivant et l’admirateur de la diversité animale. Un tel travail passe par une communication d’ampleur, menée par des professionnels appuyés par l’État, afin de recréer ces liens essentiels entre la société française et son agriculture. Il paraît donc essentiel de faire de l’avenir de l’agriculture française une grande cause nationale. Quel

régulièrement au cœur des rapports de force, à l’image de l’agriculture dans son acception large. Le rééquilibrage des priorités nationales visées par le projet de loi doit aussi concerner ces outils. En soixante dix ans, la France a perdu 90 de ses outils d’abattage. La préservation de l’élevage, matérialisée par l’attention portée au maintien du cheptel et l’annonce d’un plan Abattoirs, justifie également la préservation explicite des moyens et outils d’abattage. L’amendement

L’alimentation durable est indissociable de la sécurité alimentaire, car elle renvoie à l’ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisantes.

en présence de toutes les parties prenantes des filières d’élevage. Celles ci aboutiront à des contrats sanitaires de filière pour une meilleure performance. Par

Du fait de leurs engagements régionaux et internationaux, la France et l’ensemble des États membres de l’Union européenne sont soumis à des obligations extraterritoriales et doivent s’assurer à la fois de respecter les droits humains et de ne pas porter atteinte aux droits humains dans d’autres pays protéger les populations des violations des droits humains, notamment en s’assurant que les acteurs économiques de la chaîne alimentaire qui opèrent sur le marché international ou à l’étranger ne portent pas atteinte aux droits humains, en particulier les droits des paysans, le droit à l’alimentation des populations et les droits environnementaux participer à la réalisation des droits humains à l’échelon international en mettant en œuvre des politiques de développement et une coopération internationale conformes et adaptées. Par ailleurs, nous ne comprenons absolument pas la vision de notre rapporteur, qui, de manière antithétique, propose d’améliorer tout à la fois la compétitivité

pour soutenir les capacités exportatrices de la France nécessaires à la sécurité alimentaire mondiale. Si nous souscrivons à la nécessité que la France reste une puissance exportatrice forte sur la scène mondiale, avec des filières de renom et d’exception participant clairement à notre rayonnement à l’international et, surtout, à l’équilibrage de notre balance commerciale extérieure, nous nous interrogeons toutefois sur le fait que notre pays ait vocation à assurer la sécurité alimentaire mondiale Je crains que nous ne nous trompions ici d’objectif. Si la France doit apporter sa pierre à cet édifice de recherche de sécurité alimentaire mondiale, nous n’estimons pas pour autant qu’il faille l’inscrire en l’état dans la loi, au risque de vouloir produire toujours plus, quelles qu’en soient les conditions. Par cet amendement, nous appelons à en rester à une rédaction plus sobre et réaliste, en précisant que nos politiques publiques visent à préserver nos capacités exportatrices et à maîtriser et réduire notre dépendance aux exportations.

Si l’on inscrit dans la loi qu’il faut soutenir les capacités exportatrices de la France, dans l’objectif de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, nous ne voulons pas que cet objectif soit entendu comme une course au productivisme à tous crins. Notre amendement tend ainsi à préciser que l’objectif de soutien des capacités exportatrices de notre pays ne doit en aucun cas nuire à notre souveraineté alimentaire nationale et à l’autonomie alimentaire de nos territoires.

pour refléter l’importance de ces piliers fondamentaux de la politique environnementale. Il s’agit là, bien entendu, d’un élément central pour notre souveraineté alimentaire. En effet, lorsque nous aurons perdu l’ensemble des pollinisateurs, c’est 30 % de notre production qui disparaîtra également

l’amendement du Gouvernement prenait en compte votre proposition, puisqu’il avait pour objet d’intégrer l’ensemble des actions à conduire dans le cadre de la politique de l’alimentation tout en contribuant à un objectif plus global de souveraineté alimentaire. Cette politique a notamment pour finalité d’assurer à la population l’accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée,

contre la concurrence déloyale des produits importés moins disants d’un point de vue social, environnemental et sanitaire. Alors que les normes de production dans les pays tiers autorisent des produits interdits dans l’Union européenne – pesticides, hormones de croissance, etc. dans un contexte de hausse des importations et alors que la protection des consommateurs est essentielle, la mise en place de mesures miroirs à l’échelle européenne est plus que nécessaire. Je sais que cette nécessité fait consensus sur l’ensemble de nos travées,

respectent les normes sociales, sanitaires, environnementales et relatives au bien être animal en vigueur dans l’Union européenne. Alors que la nécessaire mise en place des mesures miroirs à l’échelle européenne annoncée par le Gouvernement ne semble pas se concrétiser,

Les biens alimentaires ne sont pas des biens comme les autres. Dans le terme « agriculture », il y a « culture », et, comme la culture, l’agriculture ne doit pas être une simple marchandise

toujours plus protectrices envers les consommateurs et préservant des modèles et des filières agricoles. Je crois, comme M. le rapporteur, que tout est dit. La rédaction issue de la commission des affaires économiques me semble à la fois opérationnelle et lisible. Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

Il s’agit de remplacer « en luttant contre la faim dans le monde » par « en contribuant à la lutte contre la faim dans le monde », considérant que la France ne peut à elle seule garantir la sécurité alimentaire mondiale et lutter contre la faim dans le monde.

de la présence des abattoirs dans nos territoires. Face à l’évolution des besoins, il est essentiel d’investir dans la rénovation et la restructuration de ces infrastructures pour qu’elles restent viables, fonctionnelles et adaptées aux défis de demain. Des

dans les territoires de polyculture élevage. Je précise que les abattoirs doivent être mono espèce ou multi espèces en fonction des élevages que l’on trouve sur les territoires. Leur rénovation est une condition de la poursuite du développement

au même titre que d’autres pans de notre économie, à la lutte contre le changement climatique et à l’atténuation de ses effets. Selon nous, cette précision, qui peut apparaître à la marge, reflète l’attitude que nous devons adopter face au changement climatique

le changement climatique ne va pas s’opérer de manière identique sur l’ensemble du territoire. Chez moi, à 850 mètres d’altitude, le changement climatique élargit les périodes de culture et améliore les stocks fourragers,

et à la nécessité de trouver des modes de production plus sobres et plus résilients face à la récurrence de la sécheresse dans nos territoires. Nous avons notamment en tête la viticulture qui, dans certains territoires, pourrait disparaître purement et simplement du fait du manque de précipitations. Nous n’oublions pas non plus l’appauvrissement de nos sols, victimes d’une agriculture trop intensive qui entraîne une chute de la biodiversité, une perte de rendement, mais également une diminution de la valeur nutritionnelle des aliments. L’ensemble de ces facteurs doit nous pousser à des efforts accrus en matière de recherche pour rendre notre agriculture plus résiliente. Quel

pas ! Je me suis trouvée aux côtés d’un arboriculteur, face à son champ : ses arbres étaient morts de soif.

marquée par la dignité de cet arboriculteur, face à la destruction totale de son outil de travail, simplement parce que l’accès à l’eau lui est interdit.

: La parole est à M. Michaël Weber. Cet amendement vise à inscrire le rôle de l’apiculture, la pollinisation entomophile, parmi les externalités positives de l’agriculture. L’apiculture assure un service de pollinisation au profit des cultures et de la flore sauvage. Sans pollinisation, 80 % des plantes cultivées en Europe ne survivraient pas.

l’horticulture, entre autres, dépendent de l’activité pollinisatrice des insectes. Celle ci est nécessaire à la survie de 84 % des plantes cultivées en Europe et améliore les rendements à l’échelle mondiale de 20 % à 30 %

du code rural et de la pêche maritime, « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Cet article répond pleinement à la préoccupation qui est exprimée

Cet amendement a pour objet de préciser et compléter les finalités de la politique menée en faveur de l’agriculture et de l’alimentation. À cette fin, il vise à citer explicitement l’objectif « d’entretien des paysages externalité incontournable au croisement de plusieurs politiques publiques incluant le tourisme, le cadre de vie et la sécurité incendie.

Mes chers collègues, en votant cet amendement, vous offrirez une visibilité nécessaire et indispensable à la problématique de l’accès raisonné à l’eau pour nos territoires agricoles en souffrance. La parole

En effet, les réseaux d’irrigation sont incontournables pour le maintien de l’agriculture et de ses externalités positives. Les territoires proches du littoral méditerranéen, par exemple, qui sont confrontés à de nombreux épisodes de sécheresse, en ont fortement besoin pour pérenniser leur agriculture, laquelle est indispensable à l’activité économique, à son développement et à la protection de l’environnement.

et de la pêche maritime des objectifs de surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique. Les dispositions de ce code s’aligneraient ainsi avec les différents plans publics, notamment avec les objectifs inscrits dans la déclinaison de la PAC

ce système de production est considéré par France Stratégie comme le plus abouti de l’agroécologie, alliant performance environnementale et économique. Les

En ce sens, l’agriculture biologique est centrale, puisqu’elle est plébiscitée par les jeunes qui souhaitent s’installer en agriculture : 30 % à 50 % des futurs agriculteurs et agricultrices

bio a fait ses preuves en matière économique et environnementale. Il a su créer son propre marché, qui atteint aujourd’hui plus de 13 milliards d’euros. S’il connaît des difficultés aujourd’hui,

Il s’agit également, dans un souci de visibilité et de cohérence avec l’alinéa 29, de réintroduire un objectif chiffré. L’objectif retenu est celui qui figure dans le programme national pour l’agriculture biologique, dit Ambition Bio

au vu de l’avancement de nos travaux et du nombre d’amendements restant encore en discussion sur ce projet de loi, en accord avec le Gouvernement et la commission des affaires économiques, nous pourrions ne pas siéger ce vendredi 7 février. Y a t il des observations ?…